Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous présenter la proposition de loi

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, chers collègues, la présentation de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, due à l'initiative de M. Jean-Pierre Sueur et des membres du groupe socialiste et républicain, est avant tout un symptôme, un symptôme, celui des dysfonctionnements de l'intercommunalité dans certains de nos départements à la suite des dernières réformes territoriales. Personne ne se préoccuperait outre mesure de rééquilibrer la composition des conseils communautaires si le fonctionnement de l'intercommunalité était toujours harmonieux et si le véritable esprit de coopération qui doit présider à ce fonctionnement n'avait pas été mis à mal par des regroupements forcés, par un agrandissement inconsidéré du périmètre de nombreux EPCI à fiscalité propre et par la multiplication des transferts de compétences obligatoires à leur profit. On n'accorderait peut-être pas non plus autant d'importance à ce que les conseillers municipaux qui ne sont pas membres de l'organe délibérant de l'EPCI auquel leur commune appartient soient correctement associés au fonctionnement quotidien de cet établissement si la plupart des leviers de décision n'avaient pas été transférés au niveau intercommunal. Cette proposition de loi soulève donc des questions auxquelles il est urgent d'apporter des réponses. Je me félicite de ce que le Président de la République, lors de son déplacement dans l'Eure, la semaine dernière, ait fait part de son esprit d'ouverture en la matière. Oui, il est temps de corriger certains effets pervers des dernières réformes territoriales, afin- je cite le Président de la République -de « remettre de la responsabilité au plus près du terrain Cette proposition de loi a un objet plus limité. Le premier objectif est d'améliorer la représentativité des conseils communautaires. Comme vous le savez, le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant des EPCI à fiscalité propre sont déterminés soit, dans les communautés de communes et d'agglomération, par accord local d'une majorité qualifiée de conseils municipaux, soit en application des règles de droit commun fixées par la loi. L'article 1 ne traite que de la répartition de droit commun. Celle-ci obéit aujourd'hui à quatre principes principes : les sièges doivent être répartis entre les communes sur une base essentiellement démographique ; toutefois, il est attribué au moins un siège à chaque commune, ce qui est la traduction du fait qu'un EPCI à fiscalité propre est un organisme de coopération entre communes communes ; aucune commune ne peut détenir à elle seule plus de la moitié des sièges, ce qui est la conséquence du principe de non-tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre ; enfin, aucune commune ne peut se voir attribuer plus de sièges qu'elle ne compte de conseillers municipaux. Des règles complexes de répartition ont été mises au point par le législateur pour concilier, autant que faire se peut, ces quatre principes. Sans entrer dans le détail, je rappellerai que ces règles aboutissent, au regard du nombre d'habitants, à une à une forte, voire très forte, surreprésentation des petites communes et qu'elles garantissent en général une représentation correcte des communes les plus peuplées. Mais elles ont tendance à pénaliser les communes de taille moyenne, qui sont parfois sous-représentées à hauteur de plus de 70 %. Pour corriger Pour corriger ces déséquilibres, les auteurs de la proposition de loi ont imaginé une méthode originale. Ils proposent d'adopter une nouvelle règle mathématique pour traduire le principe de représentation proportionnelle, règle que j'appellerai la méthode de l'arrondi à l'entier supérieur. Je vous invite à consulter le rapport écrit pour une présentation exhaustive. La méthode de l'arrondi à l'entier supérieur produit, par elle-même, de forts écarts de représentation et ne saurait être considérée comme permettant une traduction fidèle du principe de représentation proportionnelle. Toutefois, en l'espèce, les résultats obtenus doivent être comparés avec ceux de l'application de l'ensemble des règles de répartition prévues par le droit en vigueur, qui produit, comme je l'ai indiqué, de très forts écarts de représentation. Nous avons procédé à de nombreuses simulations, complétées par celles qui nous ont été fournies par l'Association des maires de France et par le Gouvernement. Il est apparu que l'article 1, dans sa version initiale, aboutissait effectivement à corriger légèrement la sous-représentation des communes moyennes, tendait à diminuer très fortement le nombre de sièges revenant aux plus grandes communes, qui se seraient ainsi trouvées fortement sous-représentées. Reims, par exemple, aurait perdu 34 sièges au sein de la communauté urbaine La commission des lois a estimé qu'une redistribution aussi massive des sièges serait à la fois inopportune et juridiquement fragile, eu égard à la jurisprudence constitutionnelle en la matière. Elle a donc apporté à l'article 1 un correctif indispensable, en combinant la nouvelle méthode de répartition avec un nouveau mode de détermination de l'effectif théorique du conseil communautaire, c'est-à-dire de l'effectif qui sert de base aux calculs de répartition. Cet effectif théorique ne dépendrait plus seulement de la population de l'EPCI, mais aussi du nombre de communes qui en sont membres. Avec ce correctif, la mise en oeuvre du dispositif de l'article 1 aboutirait à un rééquilibrage tout à fait raisonnable de la représentation des communes au sein des conseils communautaires. Les plus grandes communes conserveraient souvent le même nombre de sièges ou elles n'en perdraient que quelques-uns, les pertes les plus fortes concernant de grandes communes qui, compte tenu de la configuration de l'EPCI, sont déjà très avantagées par le droit en vigueur. Les communes moyennes les plus pénalisées par le droit en vigueur recevraient un siège de plus. Par ailleurs, la commission a voulu emprunter une autre voie pour rééquilibrer la composition des conseils communautaires, en assouplissant les règles relatives à l'accord local de répartition des sièges. Comme vous le savez, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, le régime de l'accord local a dû être revu- ce fut fait à l'initiative de nos collègues Jean-Pierre Sueur et Alain Richard. Ce régime a le mérite d'exister. Néanmoins, il est devenu tellement strict qu'il aboutit à des situations aberrantes. Alors même que le droit commun produit de très forts écarts de représentation entre les communes, les règles régissant l'accord local sont si contraignantes qu'elles rendent illégal un accord qui, pourtant, diminue dans l'ensemble les écarts de représentation Cela tient en partie au volant maximal de 25 % de sièges supplémentaires susceptibles d'être créés par accord local. La commission des lois a donc réintroduit, à l'article 1 , une disposition adoptée en octobre 2016 par le Sénat, sur votre votre initiative, madame la ministre, et celle de notre collègue Mathieu Darnaud. Cette disposition consiste à relever à 45 % la part de sièges supplémentaires pouvant être créés, dans le cas où cela s'avère nécessaire pour conclure un accord local. En tout état de cause, cet assouplissement ne pourrait conduire à répartir plus de dix sièges supplémentaires par rapport au droit en vigueur. En outre, il nous a semblé opportun et conforme à la jurisprudence constitutionnelle d'autoriser les accords locaux qui réduisent globalement les écarts de représentation, en tenant compte non seulement du nombre de communes, mais aussi de la population concernée par ces écarts, sans produire pour aucune commune prise isolément un écart excessif. Nous en reparlerons au cours de la discussion des articles. J'en viens à l'article 2, dont l'objet est de mieux associer les « simples » conseillers municipaux, ceux qui ne sont pas membres du conseil communautaire, au fonctionnement de l'intercommunalité. C'est un objectif que nous partageons tous. On observe aujourd'hui un grand nombre de démissions chez ces conseillers municipaux qui, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi NOTRe, ont parfois le sentiment que leur mandat a perdu de son sens. Nos collègues proposaient donc que, dans les EPCI à fiscalité propre comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le conseil communautaire ait l'obligation de délibérer pour définir les modalités de participation des conseillers municipaux aux commissions thématiques. La commission a estimé qu'une telle disposition aurait laissé les EPCI à fiscalité propre dans l'insécurité juridique et qu'il valait mieux, en tout état de cause, s'en remettre à la décision locale. En revanche, elle a voulu consacrer le droit d'information de tous les conseillers municipaux sur les affaires de l'EPCI et des syndicats dont leur commune est membre. Le Gouvernement a fait part de son intérêt pour cette proposition de loi ; je l'en remercie. Je sais qu'il subsiste quelques divergences d'appréciation entre nous, mais je ne doute pas qu'elles pourront être aplanies au cours de la navette parlementaire.

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie, cher Jean-Pierre Sueur, d'avoir déposé cette proposition de loi, dont le Gouvernement partage la philosophie. Vous cherchez à favoriser une représentation plus équilibrée de toutes les communes au sein de répondre à une demande formulée à plusieurs reprises sur le terrain par les élus locaux comme par les habitants, qui font état d'un besoin de sens, de responsabilité et de proximité dans l'exercice des politiques publiques, à tous les niveaux.

ne fallait « pas tout détricoter, mais permettre, de façon pragmatique, d'améliorer les choses, en aménageant ce qui ne fonctionne pas

Cette proposition de loi cherche à répondre à un problème dont nous partageons le diagnostic, celui de la juste représentation des communes- plus précisément, même si son titre ne l'indique pas, des communes intermédiaires -au sein de l'intercommunalité. Tout à fait ! Le code général des collectivités territoriales, dont l'article concerné a fait l'objet de six modifications en cinq ans, prévoit que la répartition des sièges s'effectue selon deux possibilités : l'application du droit commun ou la conclusion d'un accord local strictement encadré.

Puis, ces sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base de la population municipale. Enfin,

et une commune disposant de plus de la moitié des sièges à l'issue de cette même opération voit sa représentation réduite d'autant. Cette opération présente, il est vrai, le désavantage de surreprésenter les plus petites communes de l'EPCI,

de la répartition de droit commun des sièges selon des règles de représentation proportionnelle avec un nombre de sièges flottant qui ne permettaient pas l'élection des conseils communautaires sur une base essentiellement démographique, comme l'exige la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel. La commission des lois du Sénat, dont je salue le travail, a donc fait évoluer le texte, en modifiant le nombre de sièges par strate du tableau et en ne conservant que trois quarts des sièges. Elle a également modifié la base de calcul permettant de répartir les sièges entre chaque commune, en appliquant un quotient électoral arrondi à l'entier supérieur. Dans cette configuration,

Cet impact est intrinsèque au modèle de répartition que vous présentez, et il n'est pas possible de l'éviter. La question est donc de savoir si ces suppressions seront jugées acceptables par les communes concernées. Enfin, à quelques mois des élections municipales, il me semble inopportun de modifier les règles de droit commun d'un dispositif qui a été à maintes reprises examiné par le juge constitutionnel et que ce dernier a stabilisé. Je rappelle que les communes doivent Je rappelle que les communes doivent délibérer sur les accords locaux avant le 31 août 2019 ... J'avais proposé

Modifier les règles aujourd'hui laisserait très peu de temps, voire pas du tout, pour mettre au point les simulateurs nécessaires et préparer les négociations. Concernant le nouvel article 1 , je remercie la commission d'avoir réintroduit l'accord local auquel, vous le savez, je suis très attachée, car celui-ci permet de donner de la souplesse aux élus locaux pour rectifier la représentation entre communes dictée par le droit commun. Comme

Toutefois, cette proposition est soumise aux mêmes contraintes calendaires que celles évoquées précédemment. Pour cette raison,

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, la représentation des communes au sein des intercommunalités est très souvent un sujet irritant, qui durcit et crispe la relation entre élus d'un même territoire, alors que l'intercommunalité est un espace de coopération qui doit se construire sur l'intelligence territoriale et le consensus, à partir d'un projet de territoire partagé au service des habitants. L'irritation est montée d'un cran ces dernières années pour deux motifs : la décision rendue par le Conseil constitutionnel en 2014 à la suite du recours de la commune de Salbris, décision qui a réaffirmé le principe d'égalité devant le suffrage, impliquant une répartition des sièges dans les conseils communautaires sur des bases essentiellement démographiques, démographiques, et la loi NOTRe et la bonification budgétaire attachée à certaines catégories d'intercommunalité, qui ont conduit à la création d'intercommunalités « XXL au sein desquelles les petites communes ou les communes intermédiaires se sentent invisibles et impuissantes, cantonnées à un rôle de figurantes, alors que l'intercommunalité absorbe de plus en plus de compétences. Aussi convient-il de saluer la volonté exprimée par notre éminent collègue Jean-Pierre Sueur et les cosignataires de cette proposition de loi de tenter de répondre au malaise des communes et de résoudre

et rend très difficile l'application d'une règle universelle uniforme ressentie comme équitable par tous, dans le respect des exigences du Conseil constitutionnel.

Toutefois, si la volonté initiale des auteurs de cette proposition de loi était d'améliorer la représentation des petites communes, il s'est avéré, au regard des simulations effectuées, que la règle de répartition proposée aboutissait en réalité à écraser la représentation des communes intermédiaires. De ce fait, notre collègue rapporteur, dont je salue la qualité et l'importance du travail, a préféré proposer une autre méthode de redistribution des sièges. Pour autant, ma chère collègue, cette proposition déplace le problème sans véritablement le régler, ... Si ! ... car si elle satisfait 18 000 communes représentant 21 millions d'habitants, elle pourrait en irriter 14 000 regroupant 39 millions d'habitants. le risque d'inconstitutionnalité est réel, et sa réalisation aurait de lourdes conséquences pour les intercommunalités et les communes, contraintes de défaire et refaire douloureusement une composition du conseil communautaire qui doit être arrêtée au 31 août 2019. Aussi nous semble-t-il difficile de créer, par ce texte, un espoir de meilleure représentation qui serait mis à mal ultérieurement. Le Sénat, représentant des territoires, défend toujours avec conviction la nécessaire prise en compte de leur diversité pour garantir l'efficience de l'action publique. Cette diversité appelle un cadre législatif qui permette plus qu'il n'impose. Dans cette perspective, je salue encore une fois l'excellent travail de notre rapporteur, qui propose, à l'article 1 , des dispositions favorisant un assouplissement de l'accord local, dans l'esprit de la proposition

de loi ... Aujourd'hui, les règles relatives aux accords locaux sont tellement contraignantes et complexes que, dans la pratique, elles sont souvent impossibles à appliquer. Aussi la proposition de notre rapporteur de relever à 45 % la proportion de sièges supplémentaires susceptibles d'être créés par accord local est-elle une réponse intéressante. À notre sens, l'article 1 , conforté par l'amendement du Gouvernement visant à reculer l'échéance pour la détermination de la composition du conseil communautaire est véritablement de nature à diminuer le niveau d'irritation des communes. Enfin, l'article 2, qui tend à mieux associer les élus municipaux qui ne sont pas conseillers communautaires à l'action de l'EPCI, est aussi une réponse nécessaire pour atténuer le désenchantement des conseillers municipaux, qui ont l'impression d'être cantonnés à un rôle de figurant et de perdre le sens de leur engagement. Il convient tout autant d'impliquer étroitement tous les maires à l'action de l'EPCI, car ils resteront toujours comptables de l'efficacité de l'action publique devant leurs concitoyens. L'intercommunalité, espace de coopération, ne peut conduire et réussir son action sans y associer fortement et étroitement les maires et tous les élus. C'est par la construction collective d'un projet de territoire partagé que l'intercommunalité trouve son sens et recueille l'adhésion indispensable à son action. Vous l'aurez compris, le groupe Union Centriste, très attaché à la liberté des territoires, mais aussi à la sécurité de la loi et à la stabilité des dispositions législatives, notamment sur ces sujets, déterminera son vote en fonction de l'évolution du texte au cours de la séance.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires tend à répondre aux demandes de certains de ces élus qui considèrent que les évolutions récentes ont conduit à minorer leur représentation au sein des conseils intercommunaux. Ce texte a pour objet, dans un premier temps, de réformer les règles régissant la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant en prévoyant que celle-ci se fasse, dans le cadre du scrutin proportionnel, à l'arrondi supérieur. Ensuite, il vise à prévoir que l'organe délibérant d'une intercommunalité inscrive dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les élus municipaux d'une commune membre participent aux réunions des commissions thématiques. Relevant que les dispositions présentées soulevaient des difficultés, le rapporteur, notre collègue Maryse Carrère, a proposé à la commission des lois de les compléter. Un premier amendement tend principalement à corriger les effets excessivement redistributifs de la nouvelle méthode de répartition proposée, en l'assortissant d'un nouveau mode de détermination de l'effectif théorique du conseil communautaire. Celui-ci serait fonction non plus seulement de la population totale de l'EPCI à fiscalité propre, mais aussi du nombre de communes qui en sont membres. dispositif de l'article 1 permettrait un rééquilibrage raisonnable de la représentation des communes au sein des conseils communautaires et assurerait un équilibre territorial favorisant une vitalité de la démocratie locale. Un deuxième amendement a introduit un article 1 relatif aux accords locaux par lesquels les conseils municipaux des communes membres des communautés de communes et d'agglomération peuvent s'écarter des règles de droit commun en matière de composition des conseils communautaires. La commission des lois a d'abord choisi de relever, sous conditions, de 25 % à 45 % la proportion de sièges supplémentaires susceptibles d'être créés par accord local, sans augmentation de l'enveloppe indemnitaire. En outre, la commission a souhaité autoriser les accords locaux qui réduisent en moyenne les écarts de représentation entre communes au regard de leur démographie. Enfin, un troisième amendement vise, afin de mieux associer les conseillers municipaux qui ne sont pas membres de l'organe délibérant de l'EPCI auquel leur commune appartient au fonctionnement des instances de coopération, à leur reconnaître un droit général à l'information sur les affaires de l'intercommunalité. Cette règle s'appliquerait aussi bien dans les EPCI à fiscalité propre que dans les syndicats de communes. Ce texte appelle de ma part deux remarques et une justification. Première remarque : il est vrai que les communes moyennes sont plutôt pénalisées, surtout dans les grandes agglomérations, mais des accords locaux existants permettent déjà de rectifier la situation. Seconde remarque : alors que les intercommunalités devront définir sous quelques mois les règles de représentation valables à partir de mars 2020, ce texte pourrait susciter des recours qui aboutiraient à ce qu'il soit déclaré inconstitutionnel. En effet, à quatorze mois des prochaines élections municipales, les délais apparaissent bien trop courts. De plus, le texte qui nous est présenté ne s'accompagne d'aucune simulation. Enfin, j'affirme

Cet amendement a permis, en instituant des strates supplémentaires, de mieux représenter les communes plus importantes. De surcroît, les conseils municipaux des petites communes sont associés dès l'instant où le délégué de la commune fait le lien entre celle-ci et l'intercommunalité. En outre, dans les domaines où l'EPCI n'est compétent que pour les actions d'intérêt communautaire, ses délibérations sont rattachées à des délibérations communales.

à celle-ci devant les conseils municipaux, à leur demande. De plus, certains EPCI ont institué dans leur règlement intérieur un conseil des maires, délégué à un vice-président ; c'est le cas de la métropole européenne de Lille. C'est donc l'articulation entre le conseiller communautaire et son conseil municipal qui compte ; augmenter le nombre de conseillers ne changera rien. J'ajoute que, en fonction du cadre juridique, certaines décisions communautaires sont soumises à une délibération communale,

Saury. Madame la présidente, madame la ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui appelés à débattre de la proposition de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires ou, sans doute plus exactement, à améliorer la représentativité des conseils communautaires et à mieux associer les conseillers municipaux au fonctionnement de l'intercommunalité. C'est un sujet important, sur lequel il est indispensable de légiférer plus justement. Beaucoup de petites communes rurales de France sont directement concernées, à l'instar de villages de mon département du Loiret. Les conseils communautaires ont été créés afin d'établir une seule instance décisionnaire, représentative des conseils municipaux d'un territoire, afin d'exercer certaines compétences que les communes ne pouvaient assumer seules. À l'origine, les accords locaux permettaient aux établissements publics de coopération intercommunale de s'adapter et aux communes de faible population de bénéficier de la présence de plusieurs représentants au sein des conseils communautaires. Cette règle de la représentation démographique avait été mise en place par la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, mais c'est la loi Chevènement du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale qui avait rendu possible les accords locaux sur la répartition des sièges au sein des organes délibérants des EPCI. La loi dite RCT de réforme des collectivités territoriales de décembre 2010 maintenait la possibilité d'accords locaux et introduisait par défaut le principe de répartition des sièges à la proportionnelle au plus fort quotient. Par une décision faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité du 20 juin 2014, dite QPC Salbris, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions législatives permettant les accords locaux au nom du principe d'égalité devant le suffrage. En pratique, il a mis un terme à toute possibilité de négocier de tels accords. En voulant protéger le principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage, les Sages ont créé une situation engendrant parfois un sentiment de frustration et d'injustice chez les élus représentant les petites communes ou les communes intermédiaires des intercommunalités. Pour trouver une solution à cette situation mal vécue par les élus concernés, les sénateurs ont été à l'initiative de l'adoption de la loi n° 2015-264, qui prévoit la possibilité de négocier de nouveau des accords locaux, mais dans des conditions moins favorables et plus complexes, notamment du fait d'écarts à la proportionnelle très faibles. En l'état actuel des choses, de nombreux élus de petites communes jugent que les évolutions législatives ont conduit à minorer de manière excessive

Si les communautés de communes et d'agglomération peuvent, selon la loi, établir elles-mêmes des répartitions de sièges, force est de constater que les critères restent très contraignants. Dans l'absolu, ceux-ci sont destinés à assurer une juste représentation devant le suffrage, mais ils s'avèrent insuffisants pour assurer un fonctionnement pour assurer un fonctionnement satisfaisant pour l'ensemble des communes membres. Devant ce constat, les auteurs de la proposition de loi tentent d'assouplir les critères de composition des conseils communautaires.

égard. À cette fin, il est proposé un système de répartition des sièges fondé sur l'arrondi à l'entier supérieur du quotient électoral. Ce système, mécaniquement plus favorable aux petites et moyennes communes, permettrait d'atténuer les décalages de représentation provoqués par la proportionnelle majoritaire et renouerait, d'une certaine façon, avec l'esprit communautaire initial. Le fait que des conseils communautaires puissent voir leur nombre de sièges majoré après l'application du nouveau mode de calcul ne semble pas constituer un obstacle majeur, car des correctifs peuvent être apportés,

C'est également un moyen de donner un poids plus important à ceux qui représentent les territoires les plus fragiles que constituent généralement nos petites communes, souvent rurales. Il s'agit véritablement, à la lumière de l'expérience de quelques années de pratique communautaire, de substituer à un strict principe d'égalité démographique un autre, fondé sur l'équité et la solidarité des territoires. Ce travail s'appuyant sur des constats posés dans nos territoires, je soutiendrai cette proposition de loi.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, le dispositif de l'accord local ayant été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans nos très éminents collègues Alain Richard et Jean-Pierre Sueur avaient déposé une proposition de loi tendant à instituer un dispositif d'accord local conforme à la jurisprudence constitutionnelle. La loi ainsi votée, intégralement validée par le Conseil constitutionnel, dispose que l'accord local doit respecter un certain nombre de règles le nombre total de sièges ne peut excéder de plus de 25 % celui qui résulterait de l'application du droit commun ; la répartition des sièges doit, conformément à la jurisprudence, s'établir en fonction de la population de chaque commune ; chaque commune dispose d'au moins un siège ; aucune commune ne peut détenir plus de la moitié des sièges la part des sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la part de sa population dans la population globale des communes membres, à deux exceptions près. On voit bien la technicité d'un tel dispositif et combien le chemin est étroit que l'encadrement de ces accords est trop contraignant et qu'il assure une trop faible représentation des petites communes au sein des intercommunalités, nos collègues ont souhaité assouplir le droit en vigueur en proposant une nouvelle méthode de répartition à la proportionnelle arrondie à l'entier supérieur. La commission a souhaité compléter ce nouveau dispositif et introduit un article 1 , visant à modifier le régime actuel de l'accord local le plafond de 25 % de sièges supplémentaires à 45 % et en ajoutant de nouvelles exceptions à la règle selon laquelle aucune commune ne peut être sur-ou sous-représentée à hauteur de plus de 20 %. qui a été modifié par la commission des lois, tend à prévoir un droit général d'information pour les conseillers municipaux ne siégeant pas dans les instances intercommunales, ce qui va dans le sens d'une plus grande transparence et d'une meilleure responsabilisation des élus qui n'appartiennent pas aux exécutifs locaux. Mes chers collègues, si nous partageons comme vous la philosophie de cette proposition de loi, qui tend à une meilleure représentation des petites et moyennes communes, nous souhaitons

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi méritoire vient après toutes les tentatives visant à rendre habitable la « baraque », ni faite ni à faire, de la réforme territoriale, sous prétexte que ce qui est fait est fait et que les élus seraient las de tout changement, même bénéfique Si la loi NOTRe, en imposant des intercommunalités regroupant un minimum de 15 000 habitants, sauf dérogations, et le bouleversement des institutions régionales et départementales ont grandement aggravé la situation et contribué à la création d'intercommunalités « XXL », ce ne sont que ce ne sont que les détonateurs d'un explosif bureaucratique dont la fabrication remonte à la loi RCT du 16 décembre 2010. En rendant obligatoire, pour la première fois, la constitution d'intercommunalités déjà plus vastes que beaucoup de celles qui existaient alors, en réglant par la loi ce qui, jusque-là, relevait du contrat statutaire entre égaux, ouvrant ainsi la voie à la transformation des EPCI intercommunaux en collectivités territoriales sans nom, en préférant la proportionnelle au plus fort quotient, qui favorise les grandes communes, à toute autre règle de répartition des sièges, la loi RCT a lancé le mouvement. mouvement sanctifié par le Conseil constitutionnel, qui s'est institué constituant en confondant sciemment intercommunalités, outils des communes pour faire à plusieurs ce qu'elles ne peuvent faire seules, et collectivités territoriales. La règle de la « représentation essentiellement démographique » n'a ici aucun sens, puisque les EPCI rassemblent des communes et non des populations, puisque les membres de leurs assemblées délibérantes représentent des communes ès qualité, et non la population de celles-ci. D'où le malaise résultant de la volonté du Conseil constitutionnel de n'en tenir aucun compte et notre présence ici pour tenter de faire baisser ce malaise d'un cran. C'est une tentative de plus ; il y en aura d'autres

Je veux bien le croire et je me rallierai d'autant plus facilement à cette version que les auteurs de la proposition de loi initiale l'ont déjà fait. Cela dit, la solution proposée par la commission n'est pas la seule possible. C'est ce que montre l'amendement de notre groupe, qui nous semble avoir un double mérite : celui d'affirmer l'existence des collectivités petites et moyennes à l'intérieur de la grande et celui de la clarté.

Dans cette optique, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, l'esprit de la coopération intercommunale nécessite parfois que l'on dépasse le simple critère de la proportionnalité démographique

Cette coopération intercommunale a ainsi constitué un outil de sauvegarde des communes, qui continuent d'exister en son sein. Or communes et intercommunalité

l'ensemble des conseillers municipaux puissent être informés de ce qui se passe à l'étage intercommunal. C'est la condition pour que la démocratie intercommunale soit vraiment fonctionnelle. En ce sens, la solution

Par ailleurs, la mise en place d'un accord dit « local » permettant de corriger des écarts de représentation est soumise à des contraintes extrêmement fortes.

de l'intercommunalité est devenu inconstitutionnel, alors qu'un accord légal, qui peut aussi présenter de fortes ruptures de proportionnalité démographique, est, quant à lui, constitutionnel.

Malgré le vote de la loi de 2015, les accords locaux doivent donc être transformés.

Il nous est apparu à tous essentiel d'assurer une meilleure représentation des communes, singulièrement de celles qui sont dans un entre-deux et de desserrer l'étau de la jurisprudence constitutionnelle.

Enfin, en ce qui concerne l'article 2, mieux associer les conseillers municipaux aux décisions communautaires est une nécessité absolue si nous voulons que le couple commune-intercommunalité puisse mieux fonctionner à l'avenir. dispositif auquel nous avons abouti à l'issue des travaux de la commission est un compromis. Il représente un premier pas, il renforce l'information ; sans doute devrons-nous aller plus loin.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui répond à l'ambition de s'attaquer au problème de la représentation de certaines communes au sein des EPCI à fiscalité propre.

le fonctionnement de ces groupements de communes, un fonctionnement qui a été bien mis à mal par un agrandissement incohérent du périmètre des EPCI et un transfert de plus en plus important de compétences des communes vers l'intercommunalité. Tout d'abord, je voudrais préciser que si la loi NOTRe a incontestablement aggravé la situation, elle ne l'a pas créée : c'est la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 qui en est à l'origine. Cette loi, associée à une interprétation très contestable du Conseil constitutionnel, a transformé le statut des intercommunalités, pour en faire quasiment des collectivités territoriales. Quant à la loi NOTRe, elle a été votée sur la base d'un rapport de la commissaire à l'égalité des territoires de l'époque, préconisant de retenir un seuil minimal de 20 000 habitants pour les EPCI. On a donc créé des intercommunalités « XXL », dont les contours ne sont aucunement cohérents

Des conseils communautaires comptant 80, 100, voire 120 membres deviennent de plus en plus de véritables chambres d'enregistrement. Une fois de plus, comme avec la fusion des régions, c'est la relation de proximité

Cette proposition de loi va donc dans le bon sens. La nouvelle méthode légale de répartition proposée au travers de ce texte, notamment par le biais du dispositif de son article 1, qui fait dépendre la représentation des communes non seulement de la population de l'EPCI à fiscalité propre, mais aussi du nombre de communes membres, nous semble assurer un rééquilibrage équitable des conseils communautaires, en favorisant la représentation des moyennes communes, qui sont les grandes perdantes du système actuel. Il en est de même de l'assouplissement des règles de l'accord local. S'agissant du droit général d'information des conseillers municipaux sur les affaires intercommunales, nous pensons qu'il permettra de les associer plus étroitement qu'aujourd'hui au fonctionnement de l'intercommunalité. J'attire également l'attention sur l'amendement déposé par notre excellent collègue Jacques Mézard qui vise à aider les maires des petites communes à mieux se faire entendre au sein de l'intercommunalité. La conférence des maires permettra une meilleure coordination entre l'intercommunalité et les communes et favorisera le consensus. Je le redis, cette proposition de loi va dans le bon sens. C'est la raison pour laquelle

Les intercommunalités représentent les communes, et non leurs habitants. Il est donc nécessaire de revoir leurs compétences. Écoutons, madame la ministre, la voix des élus de nos communes et redonnons-leur du

Madame la présidente, madame la ministre,

Malheureusement, nous constatons aujourd'hui un découragement inquiétant des élus territoriaux, qui se désespèrent du transfert des compétences, de la réduction des moyens financiers et de la perte du pouvoir de décision et de discussion au sein des grandes assemblées. Les EPCI ont pris une place considérable. Si l'on peut parfois le regretter, car cela se fait au détriment des communes, nous devons, me semble-t-il, l'accepter ; il me paraît dangereux de vouloir détricoter une fois de plus un équilibre qui a été difficile à trouver. Cela étant, comme l'a souligné le Président de la République, cela ne nous empêche pas d'améliorer les choses. Je pense que la représentation des communes au sein des conseils communautaires est un sujet majeur.

vrai dire, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur les amendements, qui ont répondu à mes interrogations. Je pense en particulier à une disposition visant à réduire les écarts de représentation.

ces jeunes communautés de communes ou d'agglomération âgées d'à peine deux ou trois décennies, même si elles ne sont pas toujours bien identifiées par nos concitoyens, jouent désormais un rôle clé dans leur vie quotidienne et l'organisation de notre pays, parce qu'elles exercent de plus en plus de compétences essentielles. Les principes à la base de leur genèse sont simples et de bon sens : proximité, subsidiarité, efficacité. Un peu à l'image du rôle que joue l'Union européenne à l'égard des États qui la composent, l'intercommunalité est censée permettre de mieux faire ensemble ce que l'on peut difficilement faire seul. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », selon un proverbe africain. Néanmoins, la réussite et le bon fonctionnement d'une intercommunalité ne se décrètent pas ; ils se construisent. Il ne suffit pas d'élaborer de beaux projets de territoire, il faut aussi et surtout savoir fédérer. que chacun se sente concerné, intégré à l'aventure intercommunale, que chaque commune s'estime gagnante et que ses habitants puissent bénéficier de l'amélioration des services et des équipements permise par l'« interco ». Initialement Initialement conçue comme un outil au service des communes, l'intercommunalité n'est cependant plus toujours considérée comme telle. Parmi les causes du vague à l'âme de nombreux élus de communes moyennes ou peu peuplées,

surtout quand le maire du chef-lieu intercommunal est aussi le président de la communauté de communes ou d'agglomération. Dans l'Oise, plus de 510 des 679 communes du département comptent moins de 1 000 habitants. Le plus souvent, elles ne sont représentées que par un élu au sein de l'intercommunalité à laquelle elles appartiennent difficile, dès lors, d'y être entendues ! Au coeur de la ruralité, certains conseillers communautaires issus des communes moins peuplées se sentent ainsi vassalisés ou méprisés, et les conseils communautaires leur apparaissent comme des chambres d'enregistrement air service du nouveau marquis local. « On ne sert à rien », « tout est déjà verrouillé », entend-on souvent. Aussi, au-delà d'un juste rééquilibrage mathématique, cette proposition de loi peut aussi avoir une vertu psychologique. Il est en effet toujours préférable de se sentir considéré plutôt que mésestimé. S'il est rationnel, le critère démographique peut semer des germes de division et de tentation d'hégémonisme des grandes communes. Les accords locaux de répartition des sièges permis par la loi Chevènement de 1999 ont sans conteste été l'une des sources de l'élan intercommunal, tout comme la souplesse originelle de ces structures, leur capacité d'évoluer, leur vraie liberté politique et administrative, en termes de périmètre, de compétences, de priorités Parce que l'exercice de la démocratie intercommunale n'est pas toujours aisé, surtout lorsqu'il s'agit de faire travailler ensemble des élus issus de 40, 50, 60 ou même 90 communes, insuffler une nouvelle dynamique par une représentation plus équitable ne peut être que positif. La proposition de loi de nos collègues socialistes ainsi que les amendements de Mme le rapporteur me semblent donc appréciables, et je les voterai volontiers. Réussir l'intercommunalité, c'est rassembler des communes clans le respect de leur identité et de leur autonomie autour d'un projet de territoire. C'est l'unité dans la diversité, la solidarité pour l'efficacité

de marginaliser les communes au profit d'intercommunalités elles aussi démesurément étendues. Les parlementaires membres de la majorité du président Sarkozy, entre 2007 et 2012, et ceux appartenant à la majorité du président Hollande, entre 2012 et 2017, ont tous cautionné cette réforme très pénalisante pour les communes. Ils portent donc, les uns et les autres, une lourde responsabilité au regard des difficultés que rencontrent les communes en général, et plus particulièrement les petites communes en milieu rural. Il est quelque peu hypocrite- c'est le moins que l'on puisse dire -de proposer maintenant de petits aménagements qui ne règlent strictement rien sur le fond et qui ont essentiellement pour objet de dégager la responsabilité de ceux qui ont cautionné et voté toutes ces lois. La loi NOTRe a ainsi été adoptée à une très forte majorité par le Sénat et par l'Assemblée nationale ; il en avait été de même, à l'époque du président Sarkozy, pour les lois qui ont imposé un seuil minimum de population pour les EPCI et un redécoupage autoritaire des intercommunalités. À cela s'ajoutent des transferts massifs de compétences, qui ne tiennent pas compte des souhaits des collectivités concernées. Ainsi, il est évident que la vraie solution passe par une remise en cause globale de la réforme territoriale, et non par une petite rectification purement cosmétique. La

la réforme proposée avait pour effet de rapprocher de la moyenne, en termes de représentation, un nombre plus important de communes qu'elle n'en éloignait. Dans le cas d'espèce qui lui était soumis, les communes pour lesquelles l'écart à la moyenne diminuait étaient à la fois plus nombreuses et plus peuplées que les communes connaissant une évolution contraire.

à quelques mois des élections municipales, il ne me semble pas opportun de modifier les règles de droit commun d'un dispositif ayant été examiné à maintes reprises

aux communes les moins peuplées : mathématiquement, elles sont donc surreprésentées par rapport à leur population. Le problème que nous cherchons tous, depuis longtemps,

pour explication de vote. Madame la ministre, tout cela me fait penser à la célèbre formule du père Queuille, selon laquelle il faut faire en sorte que l'impôt rende plus sans imposer plus les contribuables

dans l'exercice de leurs compétences, mettant simplement en commun des moyens, avec des élus qui sont ceux des communes, et non pas des élus intercommunaux.

à l'état d'esprit que l'on réussit à mettre en oeuvre dans la coopération entre les représentants des communes. Ce défi est d'ailleurs parfois parfois difficile à relever, tant certaines de nos intercommunalités ont été constituées à partir d'un nombre sans doute excessif

dans les intercommunalités, en desserrant quelque peu ce carcan qui a été construit non par le législateur, mais par le juge constitutionnel, s'appuyant sur

où le constituant, au nom du peuple français, doit s'emparer de ce type de questions pour faire progresser la démocratie. Cela étant, à ce stade, nous n'allons pas adopter un texte inconstitutionnel, d'autant que nous savons que la clé du problème est dans la révision de la Constitution, et non pas dans la

de la création d'intercommunalités démesurément étendues, les conseils communautaires comportent parfois un nombre considérable de membres. Or, au-delà de 100 membres, il n'y a bien souvent pas de débat possible, les pouvoirs étant concentrés dans les mains de quelques élus qui tirent les ficelles. Au moment où l'opinion publique se plaint déjà du nombre excessif d'élus à tous les niveaux, il ne serait pas raisonnable de transformer les conseils communautaires en armées mexicaines. Dans certains cas, l'efficacité est inversement proportionnelle au nombre de délégués. Le problème actuel provient de la fusion autoritaire des intercommunalités, qui a créé des structures démesurément étendues. La solution réside dans la réduction de la taille des intercommunalités plutôt que dans la multiplication d'assemblées communautaires aux effectifs pléthoriques.

dans certains EPCI à fiscalité propre. Nous avons d'ailleurs prévu que la réforme s'opérerait à enveloppe indemnitaire constante. Lorsqu'un EPCI compte plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de communes membres, il est inévitable que son conseil communautaire soit étoffé si l'on veut que l'ensemble des communes y soit représentées.

besoin ! Quel est l'avis de la commission ?

La commission se félicite du dépôt de cet amendement, qui témoigne de la volonté du Gouvernement de faire aboutir la navette parlementaire en temps utile pour que les assouplissements que nous proposons puissent s'appliquer dès les élections municipales de 2020. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Nous proposons tout simplement de rendre obligatoire la création, dans chaque EPCI à fiscalité propre, d'une instance de dialogue réunissant tous les maires des communes membres, afin de garantir la bonne coordination des actions entre les communes et l'intercommunalité et de leur permettre de débattre de projets

qui joue un rôle important pour associer ces derniers à l'action intercommunale. Nous avons toujours considéré qu'il était préférable de s'en remettre à l'initiative locale. Cependant, un sérieux problème se pose depuis l'adoption de la loi NOTRe et la refonte de la carte intercommunale qui s'est ensuivie : un grand nombre de compétences communales ont été transférées et beaucoup de maires se plaignent de ne plus

des attentes très concrètes des maires de notre pays. La belle unanimité dont vous avez fait preuve pour adopter cette mesure, mes chers collègues, témoigne du fait que chacune et chacun

faire en sorte que ce lien démocratique reste serré. Nous avons l'occasion de le signifier d'une manière fortement symbolique,

La rédaction initiale de cet article laisse entendre que les conseillers municipaux doivent prendre l'initiative de solliciter une information. Il est préférable de prévoir que, en tout état de cause, l'information doit leur être transmise.

La moindre des choses est de tenir informés les élus municipaux des communes membres des délibérations prises par l'établissement. Quel est l'avis de la commission ? ? Cette mesure est inutile : les réunions des conseils communautaires sont publiques, et leurs délibérations sont transcrites au registre des délibérations, communicables à toute personne et obligatoirement publiées au recueil des actes administratifs, dans tous les EPCI comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Mme Claudine Kauffmann. Si la note explicative sur un projet de délibération doit être transmise, il est normal que le projet de délibération lui-même soit également transmis. Quel est l'avis de la commission ?

Il est totalement inutile d'informer les conseillers municipaux des communes membres si cette information a lieu après que la délibération a été prise. Quel est l'avis de la commission ? Avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Trop souvent, les parlementaires qui ont voté certaines lois sont frappés d'amnésie. En effet, lorsque le Gouvernement change, ils font semblant de ne pas se souvenir qu'ils ont eux-mêmes cautionné les situations qu'ils dénoncent ou qu'ils critiquent. Ainsi, en ce qui concerne l'organisation territoriale, la politique qui consiste à étrangler les communes au profit des intercommunalités a été conduite de manière continue, aussi bien par le président Sarkozy que par le président Hollande. Curieusement, actuellement, on a l'impression que tout le monde déplore la situation créée et que quasiment personne n'a voté les dispositions en cause. Le présent amendement tend à rappeler implicitement les responsabilités des uns et des autres.

Malgré toutes les raisons que nous aurions de ne pas voter ce texte, nous le voterons, car il va dans la bonne direction et apporte une amélioration aux toutes petites collectivités.

la famille Rustin : c'est elle qui a inventé les rustines. Elle avait une belle entreprise sur la Vallée du Loir, à la limite du Loir-et-Cher et de la Sarthe,

est reprise. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie mercredi 23 janvier 2019 sont consultables sur le site du Sénat. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observations d'ici à la fin de la séance.

groupe socialiste et républicain, de la proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, présentée par M. David Assouline et plusieurs de ses collègues

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, le Sénat s'est souvent illustré par le passé pour sa défense intransigeante et constante des grandes libertés de notre République. Il a su mener de justes combats, au-delà du cadre partisan, pour étendre et conforter ce qui fait la dignité de l'homme. Aujourd'hui, il revient au Sénat de dénoncer un péril mortel qui menace nos démocraties. L'un de nos plus illustres prédécesseurs sur ces travées, Victor Hugo, déclarait en 1848 : « La liberté de la presse à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. » Ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui, ceux qui fustigent l'une s'en prennent aussi à l'autre. Dans le prolongement de ce long combat, je vous propose d'apporter une pierre à cet édifice jamais achevé, en adoptant cette proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des éditeurs de presse et des agences de presse. La presse telle que nous la connaissons est en déclin continu. Elle est menacée par la violence qui veut la museler. Le dernier rapport de Reporters sans Frontières fait état, pour la seule année 2018, de la mort de 80 journalistes, 49 d'entre eux ayant été assassinés en raison de leur profession.

Ils font singulièrement écho aux agressions et aux insultes qu'ont subies, ici même en France, ces dernières semaines, des représentants de la presse, leurs auteurs ayant été encouragés par des déclarations de dirigeants politiques légitimant la haine contre les journalistes. Et je passe sur tous ces États qui interdisent tout simplement l'information libre et non faussée, jusqu'à la remettre en cause au coeur de l'Europe. En outre, il y a la situation économique de la presse.

Le chiffre d'affaires de la presse baisse ainsi de plus de 4,5 % par an, ses recettes publicitaires de 7,5 %. Rien ne semble pouvoir arrêter cette spirale mortifère. Nous en voyons les conséquences autour de nous moindre couverture des événements internationaux, fermeture de marchands de presse à un rythme soutenu, quasi-faillite de Presstalis, difficultés de l'Agence France Presse, l'AFP ... C'est toute la chaîne de production de l'information qui est fragilisée

Comment opèrent-ils ? Les résultats d'une requête sur un moteur de recherche sont accompagnés, comme vous le savez, d'un résumé de quelques lignes, éventuellement agrémenté de photos. Il en est de même pour un article partagé sur un réseau social. Or ces informations suffisent très souvent à l'internaute, qui ne va presque jamais sur le site de l'éditeur. Ces, comme il convient de désigner ces résumés, constituent une spoliation des éditeurs et des agences. Sur un marché de la publicité en ligne en France estimé à 3,5 milliards d'euros, les seuls Google et Facebook en récupèrent 2,4 milliards, sans produire la moindre ligne ou la moindre photo. Les éditeurs, pour leur part, se contentent de moins de 13 % des recettes. Cette situation n'est pas nouvelle, mais elle s'est aggravée. En 2016, j'avais déposé une proposition de loi visant à instaurer un droit voisin pour les agences de presse. Les éditeurs, à l'époque, alors un peu trop confiants en la bonne volonté des plateformes, n'avaient pas souhaité y être associés. Près de trois ans plus tard, je regrette que le texte n'ait pas alors pu être au moins examiné. Cependant, la séance de ce jour, l'accueil favorable qui a été réservé jusqu'à présent à nos propositions et les échanges très constructifs, je tiens à le souligner ici, que nous avons eus avec le ministre et ses services, montrent, je pense, que nous prenons enfin la pleine mesure des risques. Le texte que je vous propose ce jour crée un nouveau droit pour les éditeurs et les agences de presse, un droit au respect des oeuvres réalisées sous leur contrôle et leur responsabilité. Cela n'aurait jamais dû cesser d'être le cas ! Tel n'est pourtant plus le cas actuellement. Concrètement, le texte va leur conférer une capacité juridique, dite « droit voisin », dans un format qui prospère déjà pour les artistes-interprètes ou les producteurs audiovisuels. Ce droit ne se substitue pas et n'enlève rien au droit d'auteur déjà reconnu aux journalistes et aux photographes. Il le rend en réalité plus efficace et adapté au monde de l'internet. En effet, ces « droits voisins » vont permettre aux éditeurs et aux agences de presse de négocier des licences auprès des moteurs de recherche et des réseaux sociaux pour l'utilisation de leurs productions, lesquelles seront bien entendu rémunérées.

je ne m'engagerai pas sur un montant, même approximatif. Il constituera de toute façon un apport important pour la presse, bien supérieur au montant dérisoire consenti par Google il y a quelques années pour solde de tout compte. Nous n'avons pas oublié les journalistes et les photographes, en un mot les auteurs, qui devront être associés aux revenus générés. La proposition de loi s'efforce de créer un cadre efficace et pleinement opérant. C'est pourquoi nous avons retenu une solution bien connue en France, c'est-à-dire la mise en place d'une ou de plusieurs sociétés de gestion collective des droits, sur le modèle de la SACEM, la Société des Beaucoup reste à faire, et ce sera l'objet de la navette avec l'Assemblée nationale. J'attire cependant d'ores et déjà l'attention de tous sur trois points cruciaux. est la mise en place d'un rapport de force favorable aux éditeurs et aux agences de presse. Les expériences de législation nationale en Allemagne et en Espagne ont mis en évidence l'influence et le pouvoir quasi monopolistique des géants de l'internet. Même la presse allemande n'a pu faire front. Pour l'instant- je dis bien : pour l'instant -, nous ne prévoyons pas d'obligation d'adhérer à une société de gestion collective. Il pourra donc y avoir plusieurs sociétés Il pourrait de même y avoir des éditeurs ou des agences tentés de faire cavalier seul, malheureusement. Ceux-là doivent bien savoir qu'ils mineraient par là même l'efficacité de nos mesures et leur propre pouvoir de négociation. Aucune agence dans le monde, aucun éditeur, ne peut instaurer à l'heure actuelle un dialogue réellement nourri- c'est un euphémisme -avec Google ou Facebook.

Un amendement de notre collègue Pierre Ouzoulias sur l'article 3 a le mérite d'évoquer cette question si importante, même si je pense que, juridiquement, sa rédaction n'est pas consolidée. Ce sera l'occasion pour nous, et pour le ministre aussi sans doute, d'affirmer, ensemble, cette nécessité. Le Le second point, en lien avec le premier, concerne la gouvernance des sociétés de gestion. Celle-ci sera complexe, à n'en pas douter, comme le seront les discussions avec les plateformes. Il faudra veiller à assurer la représentation la plus large possible des éditeurs, dans le respect du pluralisme des opinions et des formats, une représentation à l'image de la diversité de la presse. À cet égard, l'exemple de la direction de Presstalis dans le passé, confiée à une petite minorité d'éditeurs, contrairement d'ailleurs à l'esprit coopératif de la loi Bichet, a conduit à la situation très critique que nous connaissons aujourd'hui et a suscité beaucoup de ressentiment. Cela ne doit pas se reproduire. Les sociétés de gestion doivent être la maison de tous, au service de tous. Mon dernier point concerne les modalités de répartition des revenus entre les bénéficiaires. Si je ne pense pas souhaitable de fixer des règles avant même la constitution des sociétés de gestion, je rappelle que l'objet des droits voisins, en France comme en Europe, est de protéger la presse indépendante, libre, celle

et non pas les « fermes à clics » qui, par des artifices techniques et éditoriaux, comme des titres racoleurs, sont en mesure d'attirer le plus l'attention des internautes. Nous serons très attentifs, tout comme le ministre, je crois pouvoir le dire, à la bonne mise en place de ces sociétés. Cette proposition de loi, rédigée après une large concertation avec toutes les parties prenantes, adoptée à l'unanimité par la commission de la culture, dont je salue la présidente, pourrait emprunter deux chemins.

Avec l'article 13, sur le filtrage automatique des contenus postés, il a suscité des campagnes de lobbying très intenses, qui ont d'ailleurs failli réussir, puisque le Parlement européen, à la surprise générale, a dans un premier temps, le 5 juillet dernier, repoussé le texte de sa commission, avant de l'adopter finalement le 12 septembre. Depuis cette date, des réunions entre le Parlement, le Conseil et la Commission, dites « trilogues », se tiennent pour parvenir à un accord définitif. Nous étions, je dois le dire, pleins d'espoir au moment de l'adoption du texte par la Commission mercredi 16 dans l'attente de l'ultime réunion du lundi 21 janvier. Toutefois, avant même sa tenue, onze États ont, hélas, voté contre le texte de compromis, et la réunion n'a même pas eu lieu. Je comprends que cette opposition concerne davantage l'article 13 que l'article 11,

pourra peut-être nous éclairer plus avant sur les raisons de cet échec, que nous espérons tous provisoire, et sur les perspectives dans les semaines à venir. En effet, le temps presse : les élections européennes approchent, une absence d'accord avant la fin de cette législature reporterait de plusieurs années l'adoption d'un cadre commun. Ne nous y trompons pas : derrière des arguments parfois fondés, parfois moins, les opposants à cette législation, même quand ils évoquent la liberté totale et la liberté d'expression sur le Net, font le jeu des géants de l'internet, qui pour partie tirent les ficelles et souhaitent ardemment l'échec de l'Europe sur cette question, comme sur celle de la taxation. En cas de succès, ce que nous souhaitons tous, la proposition de loi pourra servir de base à une transposition rapide de la directive avec nos collègues de l'Assemblée nationale. J'ai veillé à ce que les termes du texte soient le plus possible alignés sur ceux de la directive afin que la navette soit rapidement conclusive. Dans cette optique, le texte que je vous propose laisse donc de côté pour l'instant certains éléments cruciaux, en particulier le champ des exemptions pour les. À partir de

La future directive, si future directive il y a, comme je l'espère, comportera une définition que nous pourrons intégrer au texte au cours de la navette. Dans cette attente, il me paraissait peu productif de fragiliser la position française en cours de négociation en en élaborant une

la base d'une législation nationale, susceptible d'être mise en oeuvre rapidement. Naturellement, il faudra alors que la navette nous permette d'affiner les positions des uns et des autres et que l'Assemblée nationale puisse contribuer à la construction de cette législation, mais, sur le fond, comme le montrent tous nos débats, nous sommes tous d'accord sur le principe. Dès lors, la France s'honorerait à mettre en place un dispositif efficace, qui tienne compte des expériences allemandes et espagnoles. Je ne doute pas que, le cas échéant, d'autres pays nous rejoindraient rapidement, car la France est la France. Ce que nous sommes en train de construire, ou plutôt de « coconstruire », monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est une législation qui réaffirme le caractère essentiel pour la vitalité et la qualité du débat démocratique d'une information libre, indépendante, pluraliste et produite de manière professionnelle. Je rappelle que, contrairement à ce que l'internet a pu nous conduire à penser, l'information a un coût élevé et que la situation des éditeurs et des agences, comme celle des journalistes, et peut-être plus encore des photographes de presse, est critique. C'est également une législation pour le siècle qui vient que nous élaborons,

contre le sentiment d'impuissance qui a trop longtemps dominé. C'est donc avec enthousiasme et espoir que je vous propose d'adopter cette proposition de loi. La parole est à M. le ministre.

Ils en sont les vigies. Au cours des dernières semaines, ils ont fait l'objet, vous le savez, d'attaques répétées. Des journalistes, dans notre pays, ont été agressés ; des imprimeries ont été bloquées ; le rôle de la presse est contesté. Cette violence est tout simplement inacceptable, intolérable et inexcusable. Elle est d'autant plus inacceptable et dangereuse que, à l'heure des réseaux sociaux, nous avons plus que jamais besoin de la presse

Quand les dirigeants de la France insoumise, du Rassemblement national ou encore de Debout la France ! propagent des « infox » dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux, ils sont seuls face à leur caméra, sans personne pour les contredire. Mais quand ils les reprennent, en direct à la télévision ou à la radio, il y a une différence, et une différence de taille : en face d'eux, il y a des journalistes pour les contester, pour les corriger, pour leur dire que c'est faux, et pourquoi c'est faux. Notre premier rempart contre les fausses informations, ce sont les journalistes. S'en prendre à eux, c'est s'en prendre à tout ce que nous défendons. C'est s'en prendre à la démocratie. C'est s'en prendre à la République. C'est s'en prendre, n'ayons pas peur de le dire, à la France. Il est de la responsabilité de l'État de les protéger, de les aider à exercer leur métier, de garantir leur liberté, mais c'est aussi la responsabilité de chacune et de chacun La situation est grave : le baromètre de la confiance dans les médias, rendu public ce matin, montre que cette confiance a atteint son plus bas niveau historique. Et aucun média n'est épargné aucun média n'est épargné par la montée de la défiance. Je travaille activement à trouver des solutions pour restaurer cette confiance. L'éducation aux médias-

Le droit voisin pour les éditeurs et les agences de presse, objet de la proposition de loi que vous examinez aujourd'hui, fait partie de ces solutions. En effet, pour avoir une presse de qualité, pour que les journalistes puissent

Or le modèle économique de la presse est mis à mal par la révolution numérique. Si certains acteurs n'y ont malheureusement pas survécu, et beaucoup ont su s'adapter en investissant, en se réinventant, en adoptant des modèles économiques innovants, par la publicité et les abonnements, notamment. Pourtant, malgré ces efforts, la presse continue de jouer son avenir le développement des revenus du numérique n'a pas compensé l'effondrement de l'édition papier. Si cette compensation n'a pas eu lieu, c'est en partie parce que la valeur créée par les éditeurs et les agences de presse est accaparée par d'autres, d'autres, en particulier par les plateformes, par les agrégateurs de contenus et par les moteurs de recherche, qui réutilisent leurs contenus sans les rémunérer, alors même qu'ils génèrent d'importants revenus publicitaires. Les chiffres sont édifiants les éditeurs ne captent que 13 % de la valeur générée par le marché français des agrégateurs de contenus sur internet. 13 % ! Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter que ceux qui diffusent les contenus soient démesurément mieux rémunérés que ceux qui les créent. Non seulement c'est injuste, mais c'est un danger pour l'ensemble de la presse. À travers les éditeurs et les agences de presse, c'est toute la filière qui est touchée, des journalistes jusqu'aux kiosquiers. À terme, c'est le pluralisme qui est menacé, et tout simplement la presse elle-même. Pour remédier à cette situation, nous devons garantir un juste partage de la valeur et procéder à un rééquilibrage au profit des éditeurs et des agences de presse. Nous devons leur permettre de percevoir une rémunération pour chaque réutilisation de leurs contenus. Tel est l'objectif du droit voisin. Je défends sa création, avec engagement et détermination,

Votre proposition de loi, monsieur Assouline, reprend les positions défendues par la France dans les négociations européennes en cours. Je m'en réjouis. La France se bat depuis plusieurs années pour qu'un droit voisin pour les éditeurs et les agences de presse soit reconnu à l'échelon européen, reconnu à l'échelon européen, dans le cadre des négociations sur la directive Droit d'auteur. Nous sommes aujourd'hui dans la dernière ligne droite de cette négociation, à l'étape des trilogues, vous l'avez rappelé, monsieur Assouline, c'est-à-dire des négociations entre les États membres, la Commission européenne et le Parlement européen. Depuis mon arrivée au Gouvernement, voilà maintenant trois mois, je me suis très fortement mobilisé pour faire aboutir cette phase décisive des négociations. Ce n'est pas simple. Je me suis rendu très rapidement à Bruxelles pour rencontrer mes homologues. J'échange très régulièrement avec la Commission et les parlementaires impliqués

Je dois dire, avec beaucoup de regret, qu'une partie des États membres qui s'opposent à ce droit, même s'ils sont minoritaires, le font parce qu'ils ne souhaitent pas donner plus de moyens à la presse

en tout cas une grande victoire, parce que, sur ce sujet, face aux géants numériques, nous ne ferons le poids que si nous faisons front commun, comme vous l'avez rappelé, monsieur Assouline. Jusqu'à présent, les initiatives isolées ont échoué,

L'Allemagne, où le droit voisin a été institué en 2013, est un exemple supplémentaire : Google a refusé de négocier le versement d'un pourcentage de son chiffre d'affaires, et un bon nombre d'éditeurs allemands ont fini par lui accorder une licence gratuite. La leçon à tirer de tout cela, c'est que notre seule protection efficace et crédible, c'est l'union. Les plateformes peuvent peut-être se passer de proposer leurs services dans un ou deux pays. Elles peuvent peut-être renoncer à quelques dizaines de millions d'usagers, mais elles ne peuvent pas tourner le dos à l'Europe. Elles ne peuvent pas se départir de 700 millions d'internautes potentiels ! Google, ! Google, par la voix d'un de ses dirigeants, a évoqué l'éventualité de fermer son service Actualités en Europe si le Parlement européen consacrait le droit voisin : il s'agit d'un chantage inacceptable, en plus d'une mesure improbable. Google est un partenaire pour la France, comme le Gouvernement l'a souligné lors du sommet Choose France lundi à Versailles, mais certaines pratiques comme le lobbying massif mené à Bruxelles et dans de nombreux États membres contre la directive Droit d'auteur ne sont absolument pas acceptables. Nous l'avons dit aux dirigeants de cette entreprise. Je le leur ai dit moi-même lundi. La France ne cédera pas à ces menaces. Nous irons jusqu'au bout sur ce sujet. sur ce sujet. Mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur Assouline, j'ai eu l'occasion de vous le dire : au regard du calendrier de la négociation européenne, l'examen de votre proposition de loi

Si la création d'un droit voisin est clairement prévue par le texte européen en cours de négociation, la rédaction précise de ce texte n'est pas encore tout à fait stabilisée. Toutefois, j'ai souhaité, dans un esprit de consensus, que nous puissions travailler ensemble sur ce texte, par anticipation de celui qui pourra être adopté à l'échelon européen.

Vous avez, chacune et chacun, fait preuve d'un esprit constructif, et je vous en remercie sincèrement. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui ; c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Il faut cesser de s'opposer sur tout, quand certains sujets nous rassemblent. Il faut savoir s'affranchir des appartenances partisanes et faire prévaloir l'intérêt général. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il faut savoir débattre, trouver des points d'accord,

possible. Nous montrons que le coeur de nos préoccupations, ce qui prime sur tout le reste, c'est l'intérêt de nos concitoyens, l'intérêt du pays. Il est toujours important de le rappeler et de le démontrer. Ça l'est tout particulièrement dans le moment difficile que traverse notre pays depuis plusieurs semaines. Le texte qui vous est présenté, mesdames, messieurs les sénateurs, est très proche de l'état de la négociation européenne.

pourra servir de texte de transposition lors d'une prochaine lecture, dans le cadre d'un travail de coconstruction avec l'Assemblée nationale. Dans l'hypothèse inverse, vous l'avez indiqué, monsieur Assouline, votre texte nous aiderait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

Celle-ci vise à maîtriser la mainmise des GAFA sur les contenus produits par les journalistes, les éditeurs et les agences de presse, dont la diffusion et l'exploitation à travers les réseaux sociaux ou les agrégateurs d'informations tels que Google, font la richesse des géants du web, qui règnent désormais sans partage sur le marché de l'information en ligne. Après plusieurs tentatives, classées sans suite, en 2012 et 2018 à l'Assemblée nationale, en 2016 au Sénat, nous espérons que la présente proposition de loi rencontrera cette année Les négociations sur la directive européenne sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique battent leur plein à Bruxelles, et il serait de la plus grande utilité de transposer rapidement les articles qui seront adoptés à l'issue du trilogue en cours. Il n'est plus admissible d'autoriser le pillage des contenus par les plateformes, moteurs de recherche et agrégateurs d'informations, qui exploitent les articles, tirent profit des recettes publicitaires et captent une partie du lectorat de la presse, sans pour autant reverser le moindre centime aux créateurs de contenus. L'Union européenne reste le seul rempart de protection efficace pour éviter les effets collatéraux que l'Allemagne et l'Espagne ont connus en 2013 et en 2014, après avoir mis en place des droits voisins nationaux pour la presse. valoriser financièrement leurs productions, les éditeurs de presse ont perdu plusieurs millions d'euros supplémentaires en raison du déréférencement de leurs contenus par Google News. Cette réaction témoigne du pouvoir démesuré dont bénéficient désormais les nouveaux intermédiaires que sont Facebook et Google dans la diffusion de l'information entre journalistes et lecteurs. Ils sélectionnent librement les informations qu'ils vont mettre en avant, selon le diktat d'algorithmes opaques nourris de nombre de clics et de. Monsieur Monsieur le ministre, si nous voulons contrer efficacement cette disqualification de l'information par des acteurs extraterritoriaux, nous ne pouvons faire l'économie d'une réflexion sur le fonctionnement et la transparence des algorithmes qui référencent les articles de presse. Une autre question se pose, celle de la durée de validité des droits voisins, si nous ne voulons pas décrédibiliser la France dans les négociations en cours. Sur ce sujet, les autorités françaises maintiennent un niveau d'exigence élevé, sans pour autant verrouiller pour une durée déraisonnable l'exploitation des contenus. La durée de validité des droits voisins pour la presse, fixée initialement à cinquante ans par la présente proposition de loi, paraissait exorbitante au regard de la nature du contenu dont il est question. La commission de la culture a d'abord adopté un amendement du rapporteur visant à porter cette durée à vingt puis, alors que notre groupe proposait un an, un compromis a été trouvé sur une durée de cinq ans. Sous réserve de l'adoption de l'amendement qui en résulte, nous voterons cette proposition de loi. Nous savons tous pourtant que nous n'aurons réglé qu'une petite partie du problème. Il restera le sujet de la fiscalité, de l'optimisation, des transferts de profits d'un pays à l'autre, des paradis fiscaux ; celui des pratiques anti-commerciales, des déréférencements des produits et services des concurrents, de la restriction des accès aux données, du manque de transparence des critères de recherche

Malgré tous les efforts de la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, qu'il faut saluer, malgré le ciblage d'Amazon par Donald Trump, qui, malheureusement, semble s'inscrire dans le cadre d'une animosité personnelle envers Jeff Bezos plus que dans une réelle stratégie antitrust, nous sommes encore bien loin du compte. La Standard Oil, lorsqu'elle a été démantelée en 1911 aux États-Unis grâce à la loi antitrust de 1890, était bien moins puissante que ne le sont les GAFA aujourd'hui. Il restera enfin tout le reste, notamment les problèmes majeurs que sont la diffusion de fausses nouvelles et le pillage de nos données personnelles, dont nous sommes à la fois victimes et acteurs, en laissant faire les nouveaux maîtres du monde que sont Google, Facebook ou Apple.

pour agir, sans attendre que le format de nos pensées se limite à 280 caractères par sujet, sans attendre que la vulgarité des propos et leur « viralité » soient les seuls paramètres permettant d'intéresser les algorithmes, dont semble désormais dépendre la marche du monde. « Il n'y a que Dieu, disait Tocqueville, qui puisse sans danger être tout-puissant. » C'est pourquoi la devise de Google, claironnée par ses fondateurs- -, est une belle formule il est dommage qu'elle ne soit aujourd'hui que cela. C'est donc au législateur européen, en l'occurrence, que revient la responsabilité de contraindre ses auteurs à la respecter. Il est essentiel que la France en prenne sa part. La parole est à M. Jean-Pierre

pillés par les moteurs de recherche ou les plateformes de partage, sans que ceux-ci les rémunèrent pour leur travail de production. Cette proposition consiste donc à anticiper sur la transposition en droit français de l'article 11 de la directive sur le droit d'auteur dans le marché unique

comme cela existe déjà dans les domaines du cinéma- pour les producteurs -et de la musique- pour les artistes interprètes. En effet, les journaux et les médias rémunèrent des milliers de journalistes pour produire des articles que l'on retrouve largement diffusés par les acteurs du numérique, lesquels perçoivent les revenus publicitaires colossaux générés par ces flux. En dix ans, la presse française a perdu 2,6 milliards d'euros de recettes publicitaires, alors que, dans le même temps, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche en ont gagné 3 Il y a là un effet évident de vases communicants. Naturellement, ces mêmes acteurs disent aux médias, qui fabriquent l'information, que ces derniers obtiennent de l'audience grâce à eux. Ce n'est pas tout à fait faux : plus de 60 % des lecteurs sont des internautes. Ce sont pourtant les éditeurs et les agences de presse qui dépensent d'importantes sommes pour réaliser des reportages, alors que ce sont les géants du numérique qui encaissent les fruits de la publicité. Il y a là un déséquilibre

Françoise Férat, le Sénat avait adopté à l'unanimité un article 10 mettant en place un système de gestion des droits pour assurer une rémunération aux photographes et aux plasticiens dont les oeuvres sont reproduites par un moteur de recherche ou un site de référencement sur internet. En seconde lecture, la commission de la culture culture avait ajouté un dispositif similaire pour les agences de presse, mais ce point avait été supprimé en commission mixte paritaire, les députés invoquant un risque procédural d'inconstitutionnalité, en raison de la fameuse règle de l'entonnoir. En mai dernier, notre collègue député Patrick Mignola a fait une nouvelle tentative, avec avec une proposition de loi dans le même esprit, qui fut rejetée après avis défavorable, à l'époque, du Gouvernement. Il semble aujourd'hui que les planètes se soient alignées et que le Gouvernement, dans la perspective de l'adoption prochaine de la révision de la directive

a voté le texte à l'unanimité. Après les amendements déposés par l'auteur-rapporteur et adoptés en commission, le texte de la proposition de loi se conforme le plus précisément possible au texte de la directive en cours de validation

et que celle-ci ne sera pas modifiable lors des transpositions par les États membres. En tout état de cause, nous ne nous exonérerons pas d'un nouvel examen au Sénat lors de la transposition définitive de la directive révisée, laquelle comprend bien d'autres sujets délicats, notamment dans son article 13, qui oblige les grandes plateformes à s'assurer qu'aucun des contenus qu'elles diffusent ne viole le droit d'auteur des artistes créateurs.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, chercher une information sur internet est devenu un geste de la vie quotidienne. Pour en savoir plus sur un sujet, vous introduisez quelques mots-clés sur la page d'accueil d'un moteur de recherche et vous obtenez en quelques secondes une foultitude de résultats. Le geste est simple, la réponse est rapide et le tout est gratuit. Gratuit en apparence, seulement, car, comme vous le savez tous, rien n'est jamais véritablement gratuit. Les moteurs de recherche stockent les informations relatives à vos requêtes et à votre profil, afin d'en faire des données qui prennent, très souvent à votre insu, une valeur marchande et pour lesquelles vous n'avez d'autre rétribution que le service qui vous est prodigué. Bien sûr, ces grands opérateurs d'internet que sont les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux procèdent à d'importants investissements technologiques pour dispenser leurs services ou, pour utiliser le vocabulaire en usage aujourd'hui, leurs « solutions

laquelle a cependant une grande qualité ; elle pointe une autre dimension très importante qui entoure la question de la répartition de la valeur entre les différents acteurs de la nouvelle économie numérisée quelle est la juste rétribution dont devrait bénéficier le producteur originel de l'information qui fait l'objet d'une valorisation, plus ou moins consentie, par ces nouveaux intermédiaires commerciaux que sont devenues les grandes plateformes d'internet ? Certes, les producteurs, tout comme les utilisateurs-consommateurs, de ces informations diffusées ou relayées sur le net tirent certains avantages des solutions mises en oeuvre par ces agrégateurs des contenus qu'ils produisent produisent : visibilité et accessibilité accrues de ceux-ci, renvois vers le site du média en question, voire, parfois, création d'un fonds d'aide spécifique octroyé à certains de ces producteurs d'information,

avoir quelques doutes sur l'équité de la répartition de la valeur produite entre les utilisateurs des services concernés et les grandes plateformes du numérique, il est clair, mes chers collègues, que nous n'en avons aucun

qui a donné lieu, le 12 septembre dernier, à un vote massif du Parlement européen en sa faveur. Le texte comporte notamment un article 11, qui permet à la presse et aux agences d'être rémunérées par les moteurs de recherche et les plateformes.

La proposition de loi nationale qui nous est soumise aujourd'hui s'inscrit globalement dans l'esprit des futures dispositions européennes qui devraient être adoptées. Si j'en approuve l'esprit et l'objet, je suis également, comme membre de notre commission des affaires européennes, très soucieux d'éviter tout risque de sur-transposition, voire de mal-transposition, par anticipation, des directives européennes dans le droit national. Aussi ai-je toujours quelques réserves à l'égard de tout projet de disposition législative nationale mené non pas en amont, mais en synchronie avec une directive européenne en cours de discussion. C'est pour cette raison que je tiens ici à saluer l'auteur de cette proposition de loi, notre collègue David Assouline, pour avoir accepté d'amender son texte, afin de le rendre le plus cohérent possible avec les futures dispositions qui devraient être prochainement adoptées à l'échelle européenne. Le groupe La République En Marche votera donc en faveur de ce texte ainsi révisé. Pour autant, nous devons bien avoir conscience que celui-ci est loin de tout résoudre.

est, à mon sens, un peu trop calqué sur celui des régimes mis oeuvre au profit de tiers à la création dans les domaines de la musique, du film, de la production audiovisuelle ou du livre. Elle ne tient guère compte de la nature particulière de l'information, de sa production

hasardeuse et coûteuse. C'est la raison pour laquelle mon groupe soutiendra les amendements proposant une limitation de ces droits à une durée de cinq ans,

Au passage, je rappelle qu'il existe une commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins, qui publie chaque année un rapport, souvent assez édifiant quant au fonctionnement de certaines de ces sociétés.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre assemblée s'est saisie, en cette séance, par le biais de cette proposition de loi, d'une affaire sérieuse : une affaire de vol, une spoliation à grande échelle de productions intellectuelles, qui lèse celles et ceux qui contribuent à l'information et menace, par là même, les fondements de notre démocratie et la capacité de nos concitoyens à se forger une opinion par la confrontation de faits collectés, commentés et soumis à leur jugement, selon des règles déontologiques acceptées collectivement. Cette dépossession sans contrepartie du travail des journalistes, aux dépens des organes d'information qui les font vivre, est organisée avec une très grande efficacité par des plateformes qui exploitent l'absence de régulation de l'internet pour profiter d'une quasi-impunité. Ce larcin est à la mesure du profit qu'elles en tirent. En 2017, Facebook a réalisé un bénéfice de près de 14 milliards d'euros et Google de près de 11 milliards d'euros. Il s'agit de résultats quasiment nets, puisque ces entités déploient des stratagèmes tout aussi démoniaques pour ne pas payer l'impôt. En très peu de temps, se sont ainsi constituées des organisations supranationales qui imposent leurs choix aux États et finiront par accaparer les derniers instruments de la souveraineté : l'émission de la monnaie et le contrôle de la démocratie. Elles exercent d'ailleurs, passivement ou activement, une influence sur le cours des campagnes électorales. En s'affranchissant du pouvoir de régulation des États, elles ont réussi à leur imposer l'intangibilité de leur principe économique, qui consiste à capter une part toujours croissante de la richesse produite par la maîtrise de la collecte et de la mise à disposition des données de l'internet.

permanente, déploie une activité soutenue et constante en faveur d'une régulation raisonnée de l'internet. La présente proposition de loi, déposée par David Assouline et ses collègues, s'inscrit heureusement dans le prolongement de ce travail de fond. Son objet est précis, son champ d'application est limité, mais essentiel, et ses moyens d'action sont pragmatiques et déjà éprouvés dans d'autres domaines de la création. Au risque de désobliger l'humilité de notre collègue David Assouline, je dirai qu'elle s'impose avec l'évidence de ces lois de bon sens, dont on se demande pourquoi elles n'ont pas été votées plus tôt. L'unanimité de notre commission, que confirmeront, sans nul doute, nos votes à venir, vous oblige, monsieur le ministre, et doit vous inciter à rejoindre notre effort collectif pour donner à cette proposition de loi une issue favorable. Son objectif n'est pas de contraindre les institutions européennes, ni de se substituer à ces dernières dans une négociation qui doit nécessairement aboutir dans le cadre de l'Union européenne. Face aux désordres de l'internet et aux risques importants qui pèsent sur le pluralisme de l'information et sur l'existence des journalismes qui en sont des acteurs et les garants, nous devons réaffirmer le principe fondamental du droit de l'auteur dans toutes ses composantes morales et économiques. En France, les droits des auteurs ont été reconnus par sept lois adoptées entre 1791 et 1793. Celles-ci ont abrogé les règles d'Ancien Régime qui donnaient au seul souverain le privilège d'autoriser et de censurer les oeuvres de l'esprit. La liberté de l'auteur et la reconnaissance de sa capacité à tirer un profit matériel de son travail intellectuel sont des acquis majeurs de la Révolution et constituent des fondements essentiels de notre démocratie. Monsieur le ministre, mes chers collègues du Parlement européen, je vous invite à considérer cette proposition de loi comme la réaffirmation solennelle de ces principes fondamentaux et l'expression de notre volonté de les mettre au service de l'élaboration d'une démocratie européenne partagée, dans les frontières de l'Union. Il ne peut subsister de démocratie véritable sans liberté d'opinion, sans reconnaissance du travail de celles et ceux qui construisent l'information et sans défense des sociétés et des organismes qui la diffusent. En protégeant les producteurs de l'information, nous donnons aussi, paradoxalement, aux plateformes la possibilité d'en tirer profit durablement. En effet, comment ne pas comprendre que leurs activités prédatrices détruisent la ressource qu'elles exploitent ? Absolument ! Cet accaparement sans contrepartie est suicidaire. Que restera-t-il sur ces réseaux quand journalistes et organes d'information auront disparu ? individuels livrés, sans élaboration, sans contrôle et sans limites, à la scoptophilie ! Le consensus trouvé en commission comme, je l'espère, dans cet hémicycle nous invite à espérer que cette proposition de loi marquera la première étape du chantier de régulation de l'internet que nous appelons collectivement de nos voeux. Le Gouvernement et l'Assemblée nationale doivent maintenant y prendre toute leur part, de façon constructive, mais dans le respect des grands principes que ce texte tend à établir. La parole

madame la présidente de la commission, mes chers collègues, il y a « urgence démocratique ! » C'est par ces termes que les entreprises de presse ont évoqué, dans une tribune du 17 avril 2018, la reconnaissance de droits voisins comme condition indispensable à à la consolidation de l'avenir de la presse. Je félicite notre collègue David Assouline pour cette proposition de loi ainsi que pour sa constance dans la défense de cette question cruciale pour notre économie comme pour la qualité de l'information. Le moment est particulièrement bien choisi pour soutenir cette proposition. Depuis que nous savons que les tractations qui devaient avoir lieu il y a trois jours ont été ajournées faute d'accord, nous souhaitons renouveler notre entier soutien aux négociateurs français, afin qu'ils aboutissent à une solution communautaire, dans les derniers mois qu'il leur reste. opposant les États membres doivent se régler au plus vite, car les plateformes et autres moteurs de recherche tireraient avantageusement parti de tels désaccords au détriment, malheureusement, des agences, des éditeurs de presse et des journalistes. Si nous défendons, bien évidemment, la position française dans la négociation à Bruxelles, nous soutenons aussi la possibilité d'aboutir à une législation nationale en cas d'échec de ces négociations. Je regrette que le projet de directive ait été la cible d'une campagne de lobbying massive et parfois mensongère menée auprès de l'opinion publique et des députés européens. Ces derniers auraient reçu des milliers de mails les appelant à voter contre le texte pour « sauver internet » La directrice générale de YouTube a qualifié le projet de « liberticide », au motif qu'il imposerait aux plateformes le filtrage des contenus, ce que ne prévoit nullement la directive. Très actif également, Google s'est offert des encarts publicitaires dans de grands journaux français pour faire part du risque d'une réduction de la diversité des contenus accessibles en ligne en cas de vote de la directive, puis est passé à l'action, la semaine dernière, en tronquant les résultats des recherches, et, enfin, relaie

Ce mode de pression a également été observé lors des expériences nationales conduites en Allemagne et en Espagne, qui se sont soldées par des échecs, parce que les « infomédiaires » ont utilisé leur puissance dans un rapport de force articulé souvent autour de la menace du déréférencement. sans doute également à ces tentatives nationales une gestion collective de ces nouveaux droits voisins, afin de renforcer les éditeurs face à ces « infomédiaires » dans les négociations, ce que n'oublie pas de faire cette proposition de loi. Il est tout aussi probable que ces deux pays, isolés, n'étaient pas en mesure de peser suffisamment dans le rapport de force. C'est la raison pour laquelle nos négociateurs doivent persévérer jusqu'à ce que l'accord soit conclu au niveau européen. Il faudra sans doute y passer quelques nuits ! À l'heure de la diffusion massive des fausses nouvelles, il est essentiel de maintenir la qualité de l'information, garantie par le statut même des éditeurs et agences de presse. Or l'existence de ceux-ci est aujourd'hui gravement

Puisqu'il nous faut soutenir la capacité des éditeurs de presse à financer et à valoriser au mieux le travail journalistique, je suis également favorable à la renégociation, prévue par cette proposition de loi, de la rémunération des journalistes, pour qu'ils puissent bénéficier des versements au titre des droits voisins. Plus globalement, nous devons faire entrer les plateformes et les moteurs de recherche dans un cadre démocratique, qui suppose non seulement qu'ils consentent à l'impôt, mais aussi qu'ils assument leurs responsabilités. Nous avions défendu avec force, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2019, l'article visant à mettre en place une fiscalité effective des GAFA, adopté par notre assemblée à une Nous soutenons également la position de la France sur le projet de directive instaurant une taxe sur les services numériques, présenté par la Commission européenne, qui prévoit de taxer le chiffre d'affaires

En tant que rapporteur de la commission de la culture sur les crédits de la mission « Livre et industries culturelles » du projet de loi de finances pour 2019, j'ai défendu les avancées indéniables que la directive sur le droit d'auteur prévoit en matière de propriété intellectuelle sur internet. Il s'agit aujourd'hui pour nous, à travers le soutien que nous apportons à ce texte et aux négociations européennes, de rééquilibrer le rapport de force et le partage de la valeur en faveur des éditeurs, des agences de presse et des journalistes. Mes chers collègues, j'espère que le Sénat, dans sa grande sagesse, se prononcera en faveur de cette proposition de loi, unanimement adoptée par la commission de la culture, afin

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le monde de la presse et, à travers lui, toute la vitalité la vitalité et la qualité du débat démocratique sont plus que jamais en danger. En effet, la révolution numérique et, avec elle, les nouveaux modes de communication dont nous sommes désormais familiers ont totalement bouleversé les modèles économiques en redistribuant les cartes en faveur des géants de l'internet. Parce qu'ils sont devenus des « intermédiateurs » incontournables et monopolistiques, à défaut de régulation, les GAFAM captent aujourd'hui toute la valeur ajoutée de ce qui circule sur le web. Après des années de naïveté complaisante, le monde commence enfin à comprendre que l'écosystème de l'internet, tel qu'il s'est développé à notre insu, défiait les États nations, sapait les moyens de l'action publique par l'optimisation fiscale et menaçait nos modèles économiques, sociaux, culturels et même démocratiques. Il ne faudra donc pas s'étonner que cette perte de souveraineté et cette « ultrafinanciarisation » au profit de quelques-uns fassent le lit des inquiétudes et des populismes. À ces défis, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est temps d'apporter vraiment une réponse politique à la hauteur.

information insatisfaisante et absence de consentement valable. Mais tout cela montre que l'autorégulation des plateformes n'est pas une réponse suffisante. Aujourd'hui,

on assiste à ce paradoxe que jamais l'information, ou ce qui paraît tel, n'a été aussi abondant, alors même que nos entreprises de presse n'ont jamais été aussi paupérisées. Or, à l'évidence, la meilleure façon de combattre la déferlante des fausses informations est de veiller à la vitalité et à la lisibilité des informations à caractère professionnel.

L'économie de l'attention sur laquelle s'est construit cet écosystème fait qu'il y a un intérêt économique, une rentabilité réelle, à répandre les fausses informations et à entretenir des bulles informationnelles qui enferment

ont montré les failles morales de ces sociétés dans la gestion de nos données personnelles, ainsi que dans l'utilisation non éthique des technologies de l'intelligence artificielle. Sur ces sujets, j'ai participé, le 27 novembre dernier, à la grande commission internationale qui a réuni à Londres, sur l'initiative de la Chambre des communes, des parlementaires de onze pays, à la suite du scandale Cambridge Analytica. J'ai porté la voix de notre assemblée, qui, de très longue date, mène un combat acharné pour le respect de nos libertés individuelles, en premier lieu celle des médias et de la

Si cette proposition de loi, importante, est un signal fort et constitue le versant économique d'un début de responsabilisation des plateformes,

anticoncurrentiels portant une atteinte grave et immédiate à l'économie du secteur ou à l'intérêt des consommateurs. Cela concerne toutes les entreprises. Nous sommes aujourd'hui totalement désarmés sur ces sujets face aux géants de l'internet,

Ma seconde résolution, déposée à l'occasion du débat sur la proposition de loi relative à la lutte contre les manipulations de l'information, a été adoptée le 30 novembre dernier. Elle appelle à une réouverture de la directive E-commerce, pour instaurer, enfin,

nous en dire plus. Si je plaide, bien entendu, pour l'équité fiscale qu'a évoquée M. Malhuret, celle-ci n'est pas l'alpha et l'oméga d'une action en faveur de la souveraineté numérique, et je plaide aussi pour une régulation très offensive de l'écosystème numérique, pour un régime exigeant de protection des données,

qui menace sa nature même. Je pense que l'urgence est de sortir d'un modèle numérique qui n'est pas durable et de regarder avec intérêt les mouvements qui se dessinent aujourd'hui autour des technologies éthiques, qui d'ailleurs peuvent être un nouveau terrain de croissance industrielle pour la France et pour l'Europe.

Comment se plaindre des conséquences des réseaux sociaux et de l'impact des GAFAM sur notre démocratie, quand nous leur avons ouvert si largement les portes de l'État ? » Il est temps que nous reprenions en main notre destin numérique !

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, « la plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés est l'ouvrage, fruit de la pensée de l'écrivain. Comme il est extrêmement juste que les hommes qui cultivent le domaine de la pensée tirent quelques fruits de leur travail, il faut que, pendant toute une vie, et quelques années après leur mort,

Les avancées techniques et technologiques ont certes actualisé et affiné les enjeux, mais,, la problématique centrale reste la même. Plus que tout autre, la révolution numérique a exacerbé la tension entre respect du droit d'auteur et accès à l'information. Cet idéal d'accessibilité infinie à des contenus multiples sous-tend la philosophie originelle d'internet, pensée comme un espace complètement ouvert et déréglementé. Cette vision a instillé une culture de la gratuité et donné l'impression aux utilisateurs que tout était libre de droits. Ce phénomène a été accentué par l'effet de réseau propre au numérique. Le partage instantané et continu de connaissances ou d'actualités s'est trouvé démultiplié. Les réseaux sociaux ont même renversé le paradigme : avec l'aspiration de données personnelles toujours plus nombreuses et avec des algorithmes de plus en plus sophistiqués, ce n'est plus l'usager qui part à la recherche de l'information, mais les réseaux qui la lui apportent.

Il était donc indispensable que le législateur intervienne pour mieux réguler l'ensemble de la chaîne et afin que le partage de la plus-value tirée des contenus entre les journalistes, les photographes, les agences ou éditeurs de presse et les plateformes soit équitable. La présente proposition de loi, dont je salue participe de ce rééquilibrage global et s'inscrit dans la tradition française de défense du droit d'auteur, sans lequel les créations de l'esprit seraient limitées. Plus précisément, il s'agit d'établir un droit voisin en réponse aux pratiques courantes consistant à reproduire des articles, photos, caricatures ou vidéos publiés par des médias sans avoir l'autorisation Si ces procédés sont créateurs de richesse pour les plateformes, en particulier grâce aux, ils induisent un manque à gagner considérable pour la presse, qui, en l'état actuel du droit, est dans l'incapacité juridique d'opposer un droit à rémunération pour des contenus pourtant créés ou légalement acquis

d'un gain légitime. Or les agences et éditeurs de presse sont aujourd'hui privés de ce gain légitime et doivent faire face à une captation de la valeur dérivant de leur travail par des intermédiaires qui le mettent à disposition sur le web. Ce texte est aussi Ce texte est aussi un moyen de valoriser l'activité des médias et le métier de journaliste. À l'heure où tout le monde peut être producteur et diffuseur de contenus, sans hiérarchisation de leur pertinence, il est fondamental de mettre en lumière le rôle essentiel d'éditorialisation des titres de presse. Le rapport Franceschini, adressé au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique en février dernier, souligne que la création d'un droit voisin est « la reconnaissance [ ...] du rôle indispensable et de l'importance du métier de l'éditeur de presse pour assurer l'exercice du droit à l'information ». Il s'agit d'un enjeu démocratique d'autant plus éminent que les « infox », nous le savons, prospèrent aujourd'hui. Reconnaître ce droit implique, en aval, que les agences et éditeurs de presse se montrent plus responsables dans la qualité de l'information produite. D'aucuns ont exprimé des craintes quant à son éventuelle dégradation, une course aux clics pouvant s'engager en vue d'obtenir davantage de recettes. Il est possible de répondre que les médias d'information générale affrontent d'ores et déjà cette situation, par l'intermédiaire des, sans que le traitement de l'actualité se soit détérioré. Au contraire, nombre d'entre eux ont mis en place des modules pour combattre les contre-vérités et apporter des éléments factuels aux citoyens. Le modèle économique de la plupart des titres repose sur les abonnés, qui attendent un professionnalisme et des analyses argumentées et détaillées. Faire montre de légèreté du jour au lendemain pourrait s'avérer contreproductif. Soyons donc confiants.

fluidifie l'accès aux contenus, l'usager n'ayant plus de démarches particulières à entreprendre auprès des médias. Surtout, elle représente un poids devant les GAFAM, de nature à rééquilibrer le rapport de force et à garantir aux éditeurs et agences de presse une rémunération plus équitable. Si ceux-ci se regroupent, leur pouvoir de négociation sera plus important

nous n'abandonnons ni le secteur de la presse ni les médias traditionnels, car les pouvoirs publics n'ont pas abdiqué face à l'omnipotence des GAFAM ! L'État a un pouvoir de régulation et de protection, et la protection légitime accordée aux agences et éditeurs

des propriétés des auteurs par les directeurs de spectacles : « Ma propriété seule, comme auteur dramatique, plus sacrée que toutes les autres, car elle ne me vient de personne, n'est pas sujette à conteste, pour dol, fraude ou séduction ; l'oeuvre est sortie de mon cerveau ». Il valait

La proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse va dans le bon sens. Elle est discutée au moment où la directive européenne sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique est sur le point d'être adoptée. La phase du trilogue succédant au vote, Parlement, Commission et Conseil des ministres proposeront une version finale du texte, qui, comme vous le savez, devra faire l'objet d'un nouveau vote au Parlement européen pour être définitivement adopté, avant d'être transposé dans le droit national des États membres.

de plusieurs groupes, afin d'être au plus près de l'enjeu des négociations qui pourraient aboutir à une durée moindre. Aussi, la loi issue de nos travaux pourrait servir de fondement à la transposition de la directive européenne, ce qui permettrait, je l'espère, une mise en oeuvre rapide. pourquoi une telle préoccupation ? C'est simplement parce que les règles européennes relatives au droit d'auteur ont été pensées avant l'ère du numérique et ne sont plus adaptées. La situation est plutôt inquiétante. Aujourd'hui, Google et Facebook peuvent référencer et diffuser des articles de presse, mais aussi créer des produits comme Google News, sans rien verser aux éditeurs en retour. Cela pose problème, parce que ces entreprises sont devenues l'une des principales portes d'accès à l'information. C'est un peu comme si les radios pouvaient diffuser toute la musique qu'elles souhaitent et engranger les revenus publicitaires afférents, sans jamais rémunérer les maisons de disques, comme l'expliquait la journaliste Chloé Woitier. La production des agences de presse, qu'il s'agisse d'éléments d'information sous toutes formes, d'articles, de photographies, de vidéographies d'infographies, est reprise par les moteurs de recherche et les agrégateurs, tels qu'ils sont publiés par les éditeurs de presse qui sont les clients de ces agences. Or les agences de presse ne concèdent pas à leurs clients, les éditeurs de presse, le droit d'accepter que ces contenus soient indexés et reproduits par les acteurs du numérique.

Une interdiction pénaliserait l'audience des éditeurs de presse, donc le chiffre d'affaires des agences, lequel dépend des audiences des éditeurs. Les agences se trouvent démunies face à la puissance des géants du numérique et ne parviennent pas à défendre efficacement leurs productions sur le fondement des droits de propriété intellectuelle existants. D'une part, l'exercice du droit d'auteur implique l'obligation de rapporter la preuve de l'originalité de chacun des contenus indexés et reproduits, ce qui est extrêmement difficile dans le cadre de pillages ou de reprises massives de contenus. des bases de données requiert notamment que toutes les extractions non autorisées soient identifiées, ce qui aboutit à de très lourdes procédures. D'autre part, en admettant qu'une agence de presse ait exercé avec succès son droit d'auteur ou son droit de producteur de base de données auprès d'un moteur de recherche, elle s'exposerait à un déréférencement des contenus publiés. Ces contenus étant repris par les éditeurs de presse, cela conduirait à les priver de référencement sur internet, ce qui constituerait un suicide économique. Enfin, au vu du rapport de force disproportionné, une confrontation bilatérale entre les agences et les moteurs de recherche ne permettrait pas aux agences de faire valoir individuellement leurs droits. En revanche, un droit voisin qui viserait à établir des accords de licence entre, d'un côté, les grandes plateformes et, de l'autre, les médias,

Cette situation constitue également un enjeu démocratique important. Il faut peut-être rappeler que, en termes de capitalisation boursière, Amazon plus Apple égale le PIB de la France. Qu'adviendrait-il si la presse française était rachetée par ces géants de l'internet ? L'information serait dictée par les intérêts des entreprises américaines. Le directeur général du groupe Figaro expliquait que 92 % de la publicité sur les smartphones est captée par Google et Facebook. Rien n'est reversé aux agences et éditeurs de presse. Rien qu'en matière de publicité, la perte de revenus est considérable. l'on y ajoute le fait que le modèle économique des éditeurs de presse est mis en grande difficulté par la dissémination croissante de leur contenu sur les GAFA sans contrepartie financière, on peut tout simplement s'inquiéter de la fin des journaux et, donc, du contenu. d'un enjeu démocratique, d'un problème de justice sociale. C'est pourquoi, mes chers collègues, je voterai en faveur de cette proposition de loi, de ce texte qui a fait l'unanimité au sein de la commission de la culture ! La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission.

sur la durée de cinq années défendue par la France à Bruxelles, dans le contexte des négociations en cours sur l'article 11 du projet de directive européenne. À l'ère de l'instantanéité des échanges d'information, une durée de vingt ans serait excessive. Le projet de directive a retenu une durée de cinq années, qui correspond également à la position de la France dans la négociation. Sachant que la position du Conseil européen est de ramener la durée de ces droits à un an, nous souhaitons renforcer la position de notre pays sans la décrédibiliser, en inscrivant dès à présent une durée de validité de ces droits de cinq que la proposition de loi

que nous attendons toujours. Or nous avons découvert cette semaine que le Défenseur des droits avait eu communication de ces données avaient éclairé son rapport. Nous aurions aimé qu'elles éclairassent aussi notre activité de contrôle de l'action gouvernementale